La parole est à M. Rachid Temal, pour un rappel au règlement.

Éric Bocquet, sur l'article. On nous a répété à l'envi que la priorité, en matière de transition énergétique, devait être la rénovation des passoires thermiques, soit les quelque 7,4 millions de logements consommant plus de 300 kilowattheures par mètre carré et par an.

Après deux ans d'attente, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est transformé en prime. En réalité, le dispositif qu'on nous propose n'est rien d'autre qu'une nouvelle mesure d'économies budgétaires, puisque 800 millions d'euros seulement seront mobilisés l'an prochain au titre du CITE,

mais vous ne parlez pas du reste à charge pour l'installation d'un système d'isolation ou de chauffage, qui sera bien trop élevé pour les ménages modestes et très modestes qui auraient recours à cette aide. Dans ces conditions, il y a de fortes chances que vous ne dépensiez même pas les 800 millions d'euros que vous avez budgétés ... De plus, vous excluez du bénéfice du CITE les Français dont les

et du développement durable. Dans le cadre de la réforme du crédit d'impôt pour la transition énergétique, l'article 4 supprime la possibilité, pour les locataires et les occupants à titre gratuit, de bénéficier de ce crédit d'impôt au titre des travaux de rénovation énergétique qu'ils réalisent dans leur habitation principale. Une telle restriction risque de décourager la rénovation des logements en location, qui font pourtant l'objet d'un nombre de rénovations insuffisant. D'après une enquête de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) publiée en octobre 2018, 24 % des travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016

Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour les locataires et toute personne bénéficiant d'un droit d'usage et d'habitation, de bénéficier, toutes conditions remplies par ailleurs, du crédit d'impôt pour les dépenses éligibles qu'ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu'ils occupent.

le parc locatif privé est un angle mort de la politique publique de rénovation énergétique. De fait, les locataires du parc privé constituent 45 % des ménages exposés à la précarité ; les propriétaires occupants n'en représentent que 39 % et les locataires du parc social, 16 %. Un quart des locataires du parc privé déclarent souffrir du froid en hiver. Dès lors, il est décevant que le plan de rénovation énergétique lancé en juin 2018 par Nicolas Hulot, alors ministre de la transition écologique et solidaire, n'ait concerné, pour le parc privé, que les propriétaires occupants. En cohérence avec les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale des bâtiments et de neutralité carbone en 2050, la lutte contre la location de passoires énergétiques doit être une priorité de la réforme du CITE. Il paraît donc nécessaire d'étendre les aides à la rénovation énergétique aux propriétaires bailleurs, afin de les inciter à réaliser les travaux qui permettront à leurs locataires de voir leur facture énergétique baisser.

Les aides sont en train de changer, puisque nous avons décidé de passer d'un crédit d'impôt à une prime, en deux temps : pour la moitié des ménages, l'année prochaine, et, pour l'autre, en 2021. Le passage d'un crédit d'impôt à une prime est un progrès, puisque le premier était versé un an et demi après les travaux, quand la seconde sera versée dès

maintenu ? Il ne faut pas se tromper de cible : soit on prend des mesures de justice sociale, soit on prend des mesures écologiques. Si l'on veut être efficace écologiquement,

Ces chaudières à gaz à très haute performance énergétique ont vocation, monsieur le président, à remplacer le parc des chaudières des anciennes générations, contribuant ainsi à la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.

tant d'économies d'énergie que de réduction des émissions de CO2. Cet amendement prévoit donc de rendre éligibles au CITE les ménages à revenus intermédiaires qui remplacent une chaudière de technologie ancienne-

Cet amendement de repli prévoit un soutien au remplacement des équipements individuels de chauffage pour les ménages à revenus intermédiaires vivant en habitat collectif, en alignant le montant du CITE sur 600 euros. Le remplacement des chaudières vétustes par un équipement performant de type chaudière THPE implique le changement du conduit collectif d'évacuation des produits de combustion et, simultanément, de toutes les chaudières raccordées sur ce même conduit. La

pour la transition énergétique. L'alinéa 15 de l'article 4 impose un critère de surface minimale pour les équipements solaires thermiques. Or il est difficile de fixer une surface unique pour l'ensemble

risquerait soit d'être fixé à un niveau trop faible pour être utile, soit d'entraîner des installations surcapacitaires, répondant mal aux besoins des ménages. Enfin, la définition de critères spécifiques pour chacune des technologies relève du domaine réglementaire. Des discussions doivent donc être engagées pour définir la manière dont les différentes applications du solaire thermique peuvent être éligibles ; pour certaines typologies, un critère de surface pourra être pertinent, mais il ne saurait l'être pour

de ces paramètres. Cet amendement technique ne tend nullement à modifier l'engagement financier de l'État. Il vise seulement à laisser plus de latitude au pouvoir réglementaire pour définir les critères adéquats pour le solaire thermique.

Du fait du passage à un forfait par équipement et de la variété des surfaces, on a besoin d'intégrer un critère permettant d'exclure des équipements trop petits ou sous-dimensionnés. Cela peut être un critère d'efficacité énergétique ou de surface. Compte tenu des arguments que vous soulevez, je vous confirme qu'il y aura bien un critère minimal de surface spécifique à l'outre-mer. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet

Le présent amendement vise à augmenter le montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier un contribuable effectuant des travaux de rénovation. Pour rappel, le montant des dépenses prises en compte pour le calcul du CITE ne peut dépasser un plafond global pluriannuel, majoré en fonction des personnes à charge. Les auteurs du présent amendement proposent d'augmenter le montant de ce crédit d'impôt, vu le coût d'une rénovation globale. Ainsi, pour un logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d'impôt dont pourrait bénéficier le ménage, toutes dépenses éligibles confondues, ne pourrait excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 4 800 euros, au lieu de 2 400 euros, pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et la somme de 9 600 euros, au lieu de 4 800 euros, pour un couple soumis à imposition commune.

Lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, a été adopté un amendement du Gouvernement visant à permettre à ces ménages de bénéficier du CITE au titre des travaux d'isolation des parois opaques.

Afin d'atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit que 9,5 millions de logements soient équipés d'appareils de chauffage au bois en 2023, il sera pourtant essentiel de mobiliser l'ensemble des segments du marché. Par ailleurs, comme pour celle des granulés, encourager l'utilisation du bois-bûches est bénéfique pour la structuration de cette filière de production- bûcheronnage, débardage, transport, transformation, commerce et distribution -, qui représente aujourd'hui près de 14 000 emplois locaux. La parole

seule la production d'eau chaude sanitaire étant alors prise en compte. C'est pourtant un système performant et fiabilisé, qui permet une importante économie d'énergie. Je pense

à la chaleur solaire, qui est l'énergie la plus appréciée des Français d'après le baromètre 2019 établi par OpinionWay pour Qualit'EnR, l'association pour la qualité des énergies renouvelables. Il vise, en particulier,

que la production d'eau chaude sanitaire. Cet amendement tend à y remédier, en alignant le montant de prime pour le chauffage solaire collectif sur celui dont bénéficient les autres systèmes de chauffage.

à l'installation. Il est, par conséquent, proposé d'augmenter de 1 000 euros le montant du CITE qui sera accordé pour l'installation de ces PAC dans les logements collectifs. La géothermie de surface est adaptée à tout type de dynamique urbaine et à tout projet d'aménagement. Elle est la seule énergie renouvelable locale permanente et permettant de produire à la fois de la chaleur, du froid et du frais, de manière quasiment gratuite et sans accentuer le phénomène de création d'îlots de chaleur urbains, à l'inverse des climatiseurs conventionnels. Elle s'impose comme une solution énergétique qui répond à la problématique thermique du bâtiment. Elle présente un potentiel de développement considérable sur l'ensemble du territoire et peut être utilisée aussi bien pour les constructions neuves que pour les rénovations. Les mesures positives prises ces dernières années pour enrayer la diminution du nombre d'installations nouvelles ne suffisent pas à redynamiser le secteur. Il est donc essentiel de conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface, aussi bien dans le secteur de l'habitat individuel que dans celui du logement collectif. La parole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

Le dispositif proposé n'est pas créateur de charge au sens de l'article 40 de la Constitution puisque fondé sur des déclarations du Gouvernement. En effet, l'exposé des motifs de l'article 4 du PLF 2020- de même que l'évaluation préalable -précise : « étant donné les contraintes de financement plus fortes sur les ménages modestes, ceux-ci resteront éligibles

même avec le versement anticipé de la prime, le crédit d'impôt étant perçu après coup. Cet article ne permet donc pas de lutter efficacement contre les freins à la réhabilitation. Pour que cette prime soit la plus efficace,

(Cipac), qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d'améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles. La parole est à M. Michel Vaspart,

La prévention et l'indemnisation des catastrophes naturelles, qu'elles soient reconnues ou qu'elles soient un peu en dehors de la réglementation est un vrai sujet, qui doit s'appréhender de manière globale. Nous allons continuer à y travailler avec le Sénat et l'Assemblée nationale. À ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable

n° I-15 rectifié . Les collectivités locales sont aujourd'hui les fers de lance de la transition énergétique, notamment par le biais de la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux à l'échelle des intercommunalités. Ce dispositif doit permettre de structurer la mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique, même s'il convient de préciser que la pollution est l'affaire de tous et qu'elle ne s'arrête pas aux frontières d'un territoire. Néanmoins, le transfert de compétences opéré envers les collectivités concernées n'a été accompagné d'aucun transfert de moyens. Or, sans moyens adéquats, l'action de ces collectivités en faveur de la transition énergétique ne peut être qu'incomplète, voire réduite au statut de simple voeu pieux. De surcroît, ces collectivités se trouvent aujourd'hui confrontées aux restrictions budgétaires. Cet amendement vise donc à attribuer une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités compétentes en matière de transition énergétique. Cette proposition a déjà été adoptée au Sénat en 2016, en 2017 et en 2018. Elle est aujourd'hui soutenue par les territoires, par les structures représentatives des collectivités et par l'ensemble de nos concitoyens, soucieux que l'action publique locale ait les moyens de ses ambitions en matière de transition énergétique. La parole

notamment la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre et de 50 % de la consommation d'énergie finale et l'augmentation de 32 % de la part des énergies renouvelables.

vous transférez la compétence aux intercommunalités et vous les laissez en rade : zéro moyen ! Là n'est pas la réponse appropriée à la crise

Sans moyens, nous n'aurons que des incantations, des documents qu'une petite partie des élus lisent, qu'une petite partie des gens intéressés consultent,

L'objectif est de leur octroyer une fraction de la TICPE calculée de manière à ce que les communautés de communes perçoivent un montant de 10 euros par habitant, c'est-à-dire le montant moyen que coûte la mise en place d'un bouquet de services de mobilité- mobilité- transport à la demande, covoiturage, vélos en libre-service. La question du financement de la compétence mobilité est essentielle. Elle a été longuement débattue lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités.

de mettre fin aux zones blanches de la mobilité ne sera pas tenu. Ce dispositif a été supprimé par les députés, ce qui a provoqué l'échec de la CMP. Le Gouvernement nous indique que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les intercommunalités pourront compter sur le dynamisme de la part de TVA qui leur sera allouée en remplacement de la taxe d'habitation. Mais rien ne nous dit que ce supplément de TVA sera suffisant et stable dans le temps, ni que son versement sera corrélé à l'exercice de la compétence mobilité- il pourra être utilisé pour financer d'autres priorités. L'actualité des derniers mois a montré combien il était urgent de réduire les fractures sociales et les fractures territoriales en développant sur l'ensemble du territoire des solutions de substitution à la voiture individuelle.

Merci,

sur la base des textes présentés par le Gouvernement et adoptés, quelles que soient les variantes, par les assemblées, l'État soit au rendez-vous.

propre à faire évoluer les habitudes seront condamnés au tout-voiture si rien n'est fait pour que s'y développent des possibilités de mobilité différentes. Je mets

au titre des investissements locatifs intermédiaires, afin de rendre ceux-ci cohérents avec l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols. La construction de logements individuels a été à l'origine de 46 % des sols artificialisés entre 2006 et 2014. En effet, de tels logements sont souvent situés en périphérie alors que la construction collective est davantage réalisée en ville, sur des terrains déjà artificialisés. Je rappelle- je suis déjà intervenue vendredi sur ce sujet -que l'artificialisation

d'habitation collectifs et à supprimer ainsi une incitation fiscale à la construction d'habitations individuelles. Cette proposition est cohérente avec l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols qui figure dans le plan Biodiversité présenté par le Gouvernement en juillet 2018.

dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire [ ...]. Les modalités d'application du présent IV , notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget ». Ce dispositif d'incitation fiscale dans l'ancien destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu'ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé n'est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme Action coeur de ville. Cet amendement, déposé par notre collègue Bernard Bonne, vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d'une expérimentation, le dispositif d'incitation fiscale dans l'ancien, dit Denormandie ». La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans. Le dispositif ne serait étendu qu'aux métropoles ayant conclu une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat de type renouvellement urbain. Quel est l'avis de la

Ces amendements visent soit à restreindre, soit à réorienter les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement immobilier, notamment les dispositifs Pinel et Denormandie. Je partage

Le Gouvernement, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, a déjà recentré ce dispositif sur les zones où les besoins sont importants. Il n'est pas figé ; nous continuons à réfléchir pour l'améliorer,

ce dispositif est déjà ouvert dans les villes du plan « Action coeur de ville » et dans les communes ayant signé une convention d'opération de revitalisation du territoire. Quant au centre des métropoles, celles qui ont conclu une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat ou de renouvellement urbain (OPAH-RU),

rappeler, nous assistons tout de même à un net ralentissement des mises en chantier ? Souvenons-nous de ce qui s'est produit lorsque Mme Cosse a mis fin ou a restreint de manière assez brutale les dispositifs de défiscalisation qui existaient.

mais toute mesure brutale, à mon avis, aura exactement les mêmes conséquences qu'en 2013 et en 2014. Or, souvenez-vous, il avait fallu que le même gouvernement qui avait décidé de frapper sur la défiscalisation en matière d'immobilier mette le Pinel sur la table pour que la construction reparte. En un

C'est par le stockage supplémentaire de carbone dans les sols que nous parviendrons à compenser une partie des émissions de CO2 dans l'atmosphère c'est scientifiquement démontré. Tel est le sens de l'initiative « 4 pour 1 000 » lancée il y a quelques mois et à laquelle se sont joints nombre de pays, de laboratoires et de scientifiques du monde entier.

secrétaire d'État. Il s'agit d'accélérer la transition énergétique du transport maritime. Nous voulons, après des échanges approfondis avec la Commission européenne, garantir la compatibilité du régime d'aide avec le droit à des aides d'État. La réforme prévue au travers de cet amendement préserve l'effet utile de la mesure, augmente le suramortissement, tout en assurant sa solidité juridique.

En réalité, le rendement fut de 280 000 euros pour 2019, et, monsieur le secrétaire d'État, vos services espèrent recueillir- vous me direz si je me trompe -530 000 euros l'année suivante, soit- quel exploit ! -quelque 5 % de ce qui était initialement prévu. donc bien loin du « succès » du prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu, qui a augmenté considérablement le rendement de ce dernier. Or, faut-il le rappeler, il repose essentiellement sur les salariés. Est-il vrai, monsieur le secrétaire d'État, que, pour 2018, seulement six yachts ont été concernés ?

le prix de vente moyen d'une embarcation de 40 mètres était, il y a cinq ans, de douze millions. Les géants de plus de 100 mètres ont une valeur pouvant approcher les 200 millions d'euros.

que notre groupe approuvait, mais on l'a remplacé par un mauvais impôt : l'impôt sur la fortune immobilière, qui partait du postulat qu'il fallait taxer tout ce qui était improductif. Pour Pour amuser un peu, la galerie, on a inventé une taxe sur yachts, qui n'est évidemment pas à la hauteur de l'enjeu. Je persiste donc à dire que la question de la fiscalité sur la fortune a été très mal traitée.

Le scrutin est ouvert.

Cette filière unique au monde, qui a commencé son activité cette année, bénéficie d'un système de financement exceptionnel prévu dans le cadre de la loi sur la transition énergétique de 2015. Il est fondé, d'une part, sur une éco-construction prélevée auprès des producteurs et importateurs, et, d'autre part, sur une quote-part du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN), taxe dont s'acquittent les plaisanciers. Il s'agit ainsi de financer la déconstruction de l'important gisement historique de bateaux, c'est-à-dire le stock pour lequel les metteurs sur le marché n'existent plus, compte tenu de la durée de vie très longue des bateaux. Dans le cadre du Comité interministériel de la mer (CIMer)

Tout le budget et la montée en puissance de l'éco-organisme ont été bâtis sur ces engagements, afin de déconstruire 20 00 à 25 000 bateaux dans les cinq ans.

Il est essentiel pour la pérennité et le bon fonctionnement de la filière, d'une part, que ce seuil soit établi à hauteur de 3 %, et, d'autre part, que ces pourcentages pour les années 2021 et 2022 soient fixés dans le cadre de la loi, afin de se conformer aux engagements du Gouvernement.

Je comprends parfaitement le rapporteur général et la commission des finances, qui n'ont pas les moyens de refaire le budget de la Nation. Mais je ne comprends pas l'attitude du Gouvernement, qui fait des promesses et ne les tient pas

Plusieurs affectataires se partagent les recettes du DAFN : le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la collectivité de Corse dès lors que le navire a un port d'attache en Corse et qu'il a stationné au moins une fois en Corse au cours de l'année, l'État, la Société nationale de sauvetage en mer depuis le 1 janvier 2018 et les éco-organismes en charge de la filière de recyclage des navires depuis le 1 janvier 2019. » Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, nous discutons donc d'une affectation qui est déjà en vigueur depuis le 1 janvier 2019

L'an passé, lors de l'examen du projet de loi de finances, j'avais déposé un amendement identique à celui-ci, visant à empêcher la hausse de la taxation du gazole non routier Cet amendement n'avait pas été adopté. Cependant, quelques semaines plus tard, en raison notamment de mouvements de protestation des professionnels, le Gouvernement avait renoncé à mettre en place cette augmentation. Cette année, les arguments sont les mêmes. Outre le coût, estimé à 800 millions d'euros, qui sera supporté en grande partie par les collectivités locales, premier donneur d'ordre de ce secteur professionnel, l'argumentaire écologique pose problème. Non pas que les professionnels des travaux publics ne souhaitent pas être vertueux en remplaçant leur matériel roulant au GNR par des engins utilisant d'autres énergies. Mais, selon mes informations, il n'existe pas à l'heure actuelle d'engins de chantier électriques, ou alors leur autonomie est si faible qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en appoint des autres matériels.

demain si le GNR est de la même couleur que le gazole utilisé par les particuliers ? Pour toutes ces raisons, je demande la suppression de l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020.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

douanes met en place un taux réduit applicable à certains secteurs, à l'exclusion toutefois de la plupart des entreprises de l'activité extractive. Or aucun engin non routier reposant sur des technologies vertes n'est encore disponible sur le marché. Le secteur extractif, particulièrement dans les zones frontalières, ainsi que le long des axes maritimes, est exposé à la concurrence des carrières des pays frontaliers. L'explosion des coûts de production consécutive à la suppression du GNR accroîtra cette exposition à la concurrence frontalière, contre la logique même de l'économie circulaire. Quant à l'explosion des coûts en amont de la chaîne des matériaux et des travaux publics,

des industries extractives.

40 % du coût d'investissement dans les engins fonctionnant exclusivement au gaz ou à l'énergie électrique. En l'état, cette mesure manque son objet, à savoir pour l'essentiel les entreprises de l'industrie extractive. Rappelons que l'immense majorité des entreprises de ce secteur ne sont pas éligibles au tarif réduit. En d'autres termes, aucune compensation adaptée n'est prévue pour l'un des secteurs les plus impactés par la suppression du GNR.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

que pour les activités de manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes ; ces dernières activités bénéficieront, en outre, d'un tarif réduit de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE). Il faut noter que les députés ont intégré à ce dispositif,

La séance est reprise.

amendement tend à prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent ces pouzzolanes destinées à des applications industrielles, qui ont été omises.

pour l'industrie extractive, particulièrement pour la production de granulats. Afin de sécuriser l'environnement économique des entreprises concernées et d'alléger leurs charges fiscales, l'amendement vise à clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrière, en affirmant que seul le régime du foncier non bâti leur est appliqué. Cette disposition permet de trouver une solution de compensation à l'augmentation de la fiscalité relative au gazole non routier, qui affecte fortement ce secteur. Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, il est proposé de prélever à leur profit la taxe générale sur les activités polluantes, applicable aux matériaux d'extraction sur les recettes de l'État. La

à soumettre les carrières au régime du foncier non bâti et flèche la TGAP matériaux d'extraction vers les collectivités afin de compenser les pertes de recettes. Dans le double objectif de simplifier et sécuriser l'environnement économique des entreprises concernées et d'alléger leurs charges fiscales, il est donc proposé de clarifier le régime foncier applicable aux terrains de carrière en affirmant leur soumission au seul régime du foncier non bâti. Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales, la taxe générale

qu'ils soient automatisés, robotisés ou non, qui permettent d'améliorer les capacités écologiques des agroéquipements. En effet, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'engager dans la voie d'une production agricole plus respectueuse de l'environnement. Cela se matérialise par l'émergence de nouvelles pratiques et par l'usage d'équipements agricoles plus modernes, plus intelligents, plus connectés, limitant entre autres les doses d'intrants utilisés. La technologie peut être le nouvel allié de l'agriculture et, en ce sens, permettre de concilier productivité et écologie. Or ces technologies de pulvérisation ou de travail du sol

Le tarif réduit de TICPE applicable au GNR est supprimé progressivement. Afin d'accompagner les entreprises dans cette suppression, des contreparties sont envisagées. Pour inciter à l'achat de matériels peu ou pas polluants, cet article prévoit notamment un dispositif de suramortissement. Cependant, dans la rédaction actuelle, les entreprises industrielles ne peuvent bénéficier du dispositif. Or les secteurs industriels, principalement composés de PME, sont d'importants consommateurs de GNR pour leurs engins de manutention. Afin de ne pas fragiliser les PME industrielles qui font face à la concurrence internationale, cet amendement vise à préciser que celles-ci bénéficieront également du suramortissement pour l'achat de matériels propres.

Cette énergie n'est pas mentionnée, alors qu'elle permet de limiter les émissions de CO2 de l'ordre de 20 % et jusqu'à 80 % s'il s'agit de biogaz et qu'elle émet peu de NOx-

dans les produits peut nécessiter des investissements importants de la part des industriels qui produisent ces matières ou de ceux qui vont les utiliser. Pour ces derniers, le montant de ces investissements peut être un frein à l'utilisation de matières premières de recyclage, les MPR, dans leur chaîne de production. Le mécanisme comptable de suramortissement pour les investissements productifs liés à la transformation et l'incorporation de MPR permettrait aux entreprises de déduire 40 % de la valeur de l'investissement sur le bénéfice imposable. les entreprises bénéficieraient d'une économie d'impôt pouvant aller jusqu'à 40 % pour celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal. Un tel dispositif avait été introduit en 2015 par la loi pour la croissance, l'activité et permettait aux entreprises de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient d'un bien. Ce mécanisme permet d'accompagner les mesures du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, ainsi que de développer les investissements visant à modifier durablement les systèmes de production pour les rendre compatibles avec l'usage de matières recyclées, ou à permettre l'incorporation d'un taux de matières recyclées plus élevé, essentiel pour la création d'un véritable marché de la matière recyclée. La parole

Le présent amendement a pour objet d'instituer un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition de boîtiers de conversion dits « flexfuel ». Si certaines régions, comme les régions Hauts-de-France ou Grand Est, ont instauré des primes permettant la prise en charge de ces dépenses à hauteur de 250 à 300 euros, elles ne sont ouvertes qu'aux habitants de ces régions. Par ailleurs, bien que les boîtiers flexfuel suscitent un réel engouement, seuls 6000 d'entre eux ont été installés depuis 2018, selon le ministère de la transition écologique et solidaire. Dans ce contexte, il est nécessaire que l'État institue un dispositif de soutien national à l'acquisition des boîtiers flexfuel, au moins pour ceux qui font l'objet d'une homologation depuis l'arrêté du 30 novembre 2017. Cette aide pourrait prendre la forme d'une incitation fiscale. Elle serait de nature à favoriser l'accès à une mobilité durable et à lutter contre la précarité énergétique sur l'ensemble du territoire.

Cet amendement vise à permettre aux entités soumises à des obligations d'économies d'énergie- les obligés -de participer à la captation du carbone en finançant des opérations du carbone en finançant des opérations de reboisement ou de restauration d'espaces naturels. Optimiser la captation du CO2 par les forêts et par les sols constitue un levier majeur pour atteindre l'objectif de neutralité carbone que nous nous sommes fixé en 2050.

les Français dans l'usage multiple qu'ils peuvent faire des capacités et des ressources énergétiques. Il convient plutôt de réfléchir et d'accompagner nos concitoyens.

En 2018, le coût de cette double taxation a atteint 3,2 milliards d'euros pour le carburant, 1 milliard d'euros pour l'électricité, 200 millions d'euros pour le gaz, et tout autant pour le fioul domestique.

Cet amendement vise à supprimer la taxe spéciale sur les huiles et à la remplacer par une taxe sur l'huile de palme alimentaire, dont le montant augmenterait progressivement de 120 euros la tonne en 2021, 160 euros en 2022, à 200 euros en 2023, à 240 euros en 2024 et à 280 euros à partir de 2025. L'huile de palme est l'oléagineux le plus rentable, avec un rendement plus de huit fois supérieur à celui des autres cultures, comme l'huile de soja, de coco ou de colza. Pourtant, la production de l'huile de palme constitue un danger écologique et environnemental de très grande ampleur. L'extension des plantations de palmiers à huile est une cause majeure de déforestation et de dégradation des écosystèmes dans les pays du Sud. Les Malaisiens et les Indonésiens ont dû engager de vastes opérations de déforestation pour se lancer dans des monocultures extensives. L'Indonésie a ainsi déjà perdu 72 % de ses forêts. À l'échelle planétaire, cette déforestation n'est pas sans conséquence non plus, puisque les forêts absorbent de grandes quantités de gaz carbonique.

et du travail (Anses), les acides gras saturés sont consommés de manière excessive par la population française, contribuent au développement de l'obésité et favorisent les maladies cardio-vasculaires. En raison de leur richesse en acides gras saturés, les huiles de palme sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture. On y recourt de manière excessive dans la restauration collective et l'industrie agroalimentaire. Elles sont notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et l'alimentation salée ou sucrée à destination des enfants. L'amendement qui tend dans le sens de la préservation de la santé humaine, de la protection de l'environnement et des habitants, notamment ceux des territoires insulaires, premières victimes du changement climatique.

qui n'est pas utilisée en droit national. Cette situation est d'autant plus difficilement compréhensible que certaines activités de transport bénéficient, elles, d'une fiscalité plus favorable que les SDIS, alors même qu'elles concourent moins à l'intérêt général. Je rappelle simplement que, en 2017, les SDIS ont effectué plus de 3 millions d'interventions au titre du secours d'urgence aux personnes.

Il s'agit notamment des produits plastiques de grande consommation, des produits jetables, du matériel scolaire et de produits et matériaux divers, comme les textiles sanitaires et la vaisselle. Aujourd'hui, malgré le développement des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), 50 % des déchets

n'est donc prévue pour qu'ils se tournent vers l'économie circulaire : c'est une sorte de prime aux cancres ! Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement leurs installations, et payer la taxe générale sur les activités polluantes, ce qui a des

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique et de cesser de taxer aveuglément les gestionnaires de déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix en amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits.

Les recettes financières tirées de cette taxe pourraient également être consacrées au développement de l'économie circulaire et à l'accompagnement des politiques de réduction des déchets et d'éco-conception des entreprises. Le décret d'application de cette mesure pourrait éventuellement prévoir des exonérations permettant d'empêcher son application aux petites entreprises.

de combustibles par traitement thermique. La TGAP déchets tend à taxer les déchets en fonction du niveau de performance environnementale du mode de traitement utilisé. À cet égard, il n'y a aucune raison de distinguer les déchets dangereux de ceux qui ne le sont pas, les traitements adaptés à chaque type de déchets étant fixés par les normes prévues dans le code de l'environnement. Les tarifs de la TGAP déchets et ses exemptions sont appliqués sans préjudice du droit environnemental relatif au traitement des déchets. Dans ce cadre, le présent amendement vise à aligner le régime des exemptions concernant les déchets dangereux sur celui qui a trait aux déchets non dangereux.

relatif aux incinérateurs, et sans préjudice des sanctions qui existent pour les réceptions de déchets dangereux préparés dans une installation autorisée, prévue à cet effet, sous la forme de combustibles solides de récupération. En effet, seule la réception de déchets non dangereux est réglementairement permise,

Par ailleurs, le droit actuel prévoit une exemption de la TGAP déchets en cas de valorisation matière et de co-incinération Afin d'assurer la neutralité de la taxe à l'égard des différents circuits et technologies, le présent amendement vise à étendre cette exemption de traitement thermique des déchets en vue de fabriquer des combustibles, qui ne seront plus considérés comme des déchets ou une co-incinération, lorsque ce traitement ne relève ni de la valorisation matière ni de la co-incinération.

à un engagement du programme présidentiel du candidat Emmanuel Macron, qui visait à favoriser l'économie circulaire. Ainsi, la loi de finances pour 2019 a prévu un signal prix fort, en augmentant significativement, par palier, le coût de la mise en décharge et de l'incinération. Le présent amendement tend à procéder à un ajustement technique. Il s'agit d'aligner les exonérations de TGAP s'appliquant sur les déchets dangereux et les déchets non dangereux, sans changer le cas

TGAP déchets aux réceptions de déchets en vue de la fabrication de combustible par traitement thermique- incinération, pyrolyse ou gazéification -, ce qui permet, soit de valoriser l'énergie produite lors du traitement des déchets, soit de créer,

Il a donné lieu à de nombreux contrôles de l'administration douanière et à de nombreux contentieux devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Cette insécurité juridique peut conduire à des inégalités dans les rapports concurrentiels entre les acteurs du secteur,

190 sont concernés par la responsabilité élargie du producteur et, donc, sous la responsabilité d'un éco-organisme chargé de les détourner de l'élimination ; 194 kilogrammes sont des biodéchets- déchets alimentaires et déchets verts -que les collectivités sont en charge de valoriser les 184 kilogrammes restants ne disposent d'aucune filière de recyclage et sont donc nécessairement éliminés dans des installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l'élimination de ces déchets. Pourtant, elles n'ont aucune prise, ni sur la conception de ces produits sans filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il est donc injuste de les taxer pour l'élimination de ces déchets, pour lesquels il n'existe aucune solution de substitution. Le présent amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables. Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe, puisque les assujettis resteraient les exploitants, cette mesure est facile à mettre en oeuvre pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l'élimination des déchets, qui justifie l'augmentation de TGAP en discussion dans ce projet de loi de finances. En effet, avec cette mesure, l'élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manoeuvre. Nous proposons donc une fiscalité incitative

L'objectif est d'instaurer cette réfaction sous forme d'un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient assujetties à la TGAP et n'auraient pas à distinguer les taux appliqués entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l'impact sur les finances publiques à hauteur de 100 millions d'euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l'objectif de division par deux du stockage prévu par la loi. Quel est l'avis de la commission

monsieur le président.

que nous soyons moins vertueux que les départements de l'Hexagone ... Nous sommes simplement moins avancés et équipés, les filières sont moins organisées et, de ce fait, les montants pratiqués deviennent, si j'ose dire, contreproductifs.

en ressources. Le paiement de cette taxe s'effectuerait en fonction du nombre d'unités importées ou vendues aux entreprises par les grossistes et s'élèverait à 5 centimes d'euro par unité.

et sont peu recyclés, voire pas du tout. La forte production d'objets promotionnels à bas coût participe ainsi à l'épuisement des ressources. La récente polémique autour des 13 millions de distribués en 2019 lors du Tour de France démontre que cette pratique est de plus en plus mal perçue par les citoyens. Des solutions de rechange plus vertueuses et aux impacts moindres pour l'environnement existent pour les entreprises et organisations désireuses de faire la promotion de leur marque. De manière générale, alors que nous déplorons le trop-plein d'objets inutiles, ces objets sont en pleine progression. Très souvent, ils proviennent de pays asiatiques. Les externalités qui leur sont associées,